je voulais confirmer la demande de la commission des finances, déjà annoncée par son président hier, d'examiner les articles de la première partie de la façon suivante : dès maintenant l'article 1, puis les articles 9 à 15, hormis l'article 13 à à l'ouverture de la séance demain matin, les articles 2 à 5, hormis l'article 4 ; à l'ouverture de la séance du lundi 25 novembre après-midi, les articles 4, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 28, 32 et 33. Il s'agira de débattre de manière spécifique de la fiscalité énergétique et environnementale. Les autres articles seraient examinés dans l'ordre normal du dérouleur. Cette demande de priorité et de réserve inclut les amendements portant articles additionnels liés aux articles mentionnés. Je suis donc Je suis donc saisi par la commission d'une demande : tendant à examiner l'article 1, ainsi que les articles 9 à 15, sauf l'article 13, en priorité au début de cette séance tendant à réserver l'examen des articles 2 à 5, sauf l'article 4, jusqu'au début de la séance du samedi 23 novembre matin ; tendant à réserver jusqu'au début de la séance du lundi 25 novembre après-midi l'examen des articles 4, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 28, 32 et 33. Cette demande s'entend des articles et des amendements portant articles additionnels leur étant rattachés. Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité et de réserve ? Avis favorable.

Lavarde. Nous commençons là par un sujet un peu technique. Le code général des impôts prévoit un report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel. Ce report d'imposition favorise notamment la création de start-up. Cependant, le texte actuel n'a pas prévu le cas de dépôt de bilan de l'entreprise bénéficiaire de l'apport de biens immatériels avant la fin du délai de report. La plus-value devient alors immédiatement exigible. Cet amendement de ma collègue Laure Darcos a pour but de supprimer le cas de dépôt de bilan des cas prévus pour mettre un terme au report d'imposition.

Concrètement, il s'agit à la fois de porter à 22 % le taux normal de la TVA, contre 20 % actuellement, et de baisser de 0,5 point le taux de la CSG activité et de 1 point celui de la CSG remplacement. Cette mesure devrait contribuer à l'allégement du déficit public en augmentant les recettes de l'État, un objectif auquel, je crois, bon nombre d'entre nous sur ces travées sont attachés. Voilà une mesure concrète qui matérialisera les bonnes intentions proclamées à juste titre dans les discours. Au-delà du seul aspect comptable, cette mesure, très largement défendue par les membres de mon groupe, contribuera à modifier la façon dont notre pays impose les facteurs de production. En effet, si la France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires, c'est par une fiscalité qui porte surtout sur le travail et le capital, plutôt que sur la consommation. La mesure que nous vous proposons marquera un premier pas vers un basculement plus large en direction d'un système où le travail et le capital seront mieux rémunérés, et la consommation plus taxée : un choix responsable de développement durable

immédiatement du pouvoir d'achat, parce que la baisse de la CSG se voit tout de suite sur les feuilles de paie, et l'augmentation de la TVA n'est pas forcément répercutée sur tous les produits.

à 150 euros par mois, soit 14 % du budget des 80 % de retraités percevant moins de 1 000 euros par mois. Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 a instauré ce taux réduit de TVA pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections absorbantes pour les personnes incontinentes, en particulier les personnes âgées. Je rappelle que certains produits pour l'incontinence strictement masculine, tels que les étuis péniens, bénéficient déjà de ce taux réduit. Le remboursement de ces produits de première nécessité répond à un enjeu sanitaire. À défaut de pouvoir y accéder, il peut en résulter des risques d'infection grave avec des conséquences psychologiques importantes,

pas le cas. Je précise qu'une partie importante de l'approvisionnement de ces produits s'opère par voie d'appel d'offres, lancé par des groupements d'achats interhospitaliers. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement

termes de santé publique est indéniable. Cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale. C'est pourquoi je vous invite, mes chers

Mme Préville. ou de réparation, ainsi que pour l'ensemble des activités de réparation, afin de faire diminuer leur coût et d'inciter le consommateur à utiliser ces services. Il s'agit de favoriser l'allongement de la durée de vie des produits, qui doit être l'un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique. C'est un sujet d'importance propre à accompagner les changements nécessaires et vertueux que notre société se doit d'opérer. Il s'agit ni plus ni moins de favoriser le réemploi et la réparation, de réduire notre impact environnemental, d'arrêter le gâchis des ressources, et de diminuer le dont nous ne savons plus que faire. C'est un petit coup de pouce que je vous propose, bien loin de la démarche qu'il nous faudrait enclencher. L'amendement

Ce chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût qui représente, pour de nombreux ménages, une opportunité de réduire leur facture énergétique. Par ailleurs, selon le Syndicat des énergies renouvelables, le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français, notamment en milieu rural où il constitue un moyen de chauffage traditionnel, comme vous le savez. Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final.

des marchés informels vers le marché formel, pour le plus grand bénéfice des recettes de l'État et de la qualité de l'air.

La fourniture de chaleur, lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d'énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la directive européenne du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique, ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid. Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d'éviter l'utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l'habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le sud de la France, où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants,

un triplement de la consommation d'énergie pour la climatisation au niveau mondial d'ici à 2050. Le développement de l'air conditionné dans les pays émergents devrait provoquer une hausse de 50 % des émissions de CO2 d'ici à 2050. Nous devons agir, et c'est un levier que nous pouvons actionner aujourd'hui. Je mets aux voix

leur première course ou leur première compétition. De fait, même s'ils sont élevés dans l'objectif de devenir des chevaux de course ou de sport, il s'agit bien d'élevage pour ces animaux. Ils ne permettent aucun gain à leur propriétaire tant qu'ils n'ont pas effectué une première course ou une première compétition. Par ailleurs, une proportion importante des chevaux n'est finalement pas envoyée dans le circuit des courses ou du sport. Il n'y a pas de raison d'appliquer un taux plein sur des animaux d'élevage

le transport de voyageurs se voit appliquer un taux intermédiaire de 10 %. Ce taux s'applique quel que soit le mode de transport utilisé, en particulier à tous les transports en commun effectués par la route, par le rail ou par les voies aériennes ou fluviales, ou encore aux taxis et aux remontées mécaniques. À l'heure de la recherche de solutions alternatives aux véhicules individuels et de mobilités plus durables, l'accès aux transports collectifs doit plus que jamais une priorité. Cela nécessite des investissements importants de la part des acteurs privés et publics, qu'il convient d'encourager dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Tel est l'objet de cet amendement. amendement vise à rétablir l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux transports publics réguliers urbains et interurbains qui prévalait avant l'application à partir de 2012 du taux intermédiaire de 7 %, et l'augmentation de celui-ci à 10 % en 2014. Par la gauche ! Cet abaissement de taux de TVA fait partie des préconisations du récent rapport présenté au Sénat sur la gratuité des transports.

il s'agit de dire tout notre attachement au développement des transports publics, qui sont absolument essentiels, à la fois dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la cohésion sociale et notre vie collective. Il arrive

à 10 % en 2014. Cette baisse du taux de TVA permettrait d'accroître la capacité financière des autorités organisatrices de mobilité, qui auront un montant moins important à reverser à l'État sur le prix des billets, billets, et ainsi de dégager des ressources financières leur permettant d'investir dans le réseau des transports en commun et dans la qualité du service, ce qui est absolument nécessaire actuellement. La baisse de ce taux permettrait de réduire le coût du transport collectif pour les usagers, contribuant ainsi à améliorer le pouvoir d'achat des Français. Une telle mesure est déjà mise en oeuvre dans de nombreux pays européens tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège ou le Portugal, où les transports publics sont considérés comme des services de première nécessité. L'amendement

intérieure sur les produits énergétiques, ou TICPE, pour les seuls paquebots de croisière, dont on parle beaucoup ces derniers temps, à l'exception des navires utilisés pour les besoins des autorités publiques, comme le précise déjà l'article 265 du code des douanes. Ces paquebots représentent en effet une grave nuisance environnementale et sanitaire, comme en témoigne la situation de Venise, qui s'enfonce sous les eaux. Selon un rapport publié en juin par l'ONG Transport et environnement, le leader mondial de la croisière de luxe émettrait ainsi, à lui seul, plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des véhicules du continent. En mer, les teneurs en soufre admises sont jusqu'à 1 500 fois plus élevées que celles autorisées pour le diesel des voitures- 1,5 % contre 0,001 %. Compte tenu des incidences sur la santé des populations riveraines des ports maritimes qui accueillent les escales, et dans l'attente de mesures plus ambitieuses, comme l'interdiction de certains types de bateaux, le présent amendement vise à soumettre le carburant des navires concernés à la TICPE.

pour favoriser les navires de croisière les plus vertueux. Je rappelle que, par définition, un port est une infrastructure reliant différents pays.

Le Gouvernement et l'État sont aujourd'hui incapables de financer les transports publics. Ils viennent de le démontrer pour l'Île-de-France, en décidant, par exemple, pour le déploiement du Grand

voulons améliorer cette qualité, il faut bien dégager des moyens. Là encore, je rejoins Roger Karoutchi : le problème se pose de savoir où trouver les moyens pour améliorer la qualité des transports publics. Faire baisser la TVA, c'est très bien. Mais la conséquence, c'est que les recettes de l'État vont baisser

nous de rétablir le principe pollueur-payeur et de supprimer une exonération superflue dans un contexte de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. J'ai entendu que des ports-

et, malheureusement, très éloignée de nos identités et de nos préoccupations singulières. La Martinique compte énormément sur le tourisme de croisière. Environ 500 000 touristes nous visitent ainsi chaque année,

afin d'empêcher l'optimisation fiscale pratiquée par certains opérateurs de communications électroniques et fournisseurs de services de télévision. Cette pratique consiste à gonfler le chiffre d'affaires hors taxes par l'adossement aux offres assujetties au taux normal de TVA de 20 % d'un ou plusieurs services soumis à un taux réduit. Ce faisant, ces entreprises minimisent la TVA reversée à l'État, pour qui la perte de recettes est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Le dispositif en vigueur visant le seul adossement de services de presse en ligne, certains opérateurs de communications électroniques et fournisseurs de services de télévision associent désormais à leurs offres des catalogues de livres en ligne, ou, et d'abonnement de cinéma, soumis au taux de 5,5 %. Il conviendrait donc d'étendre le dispositif adopté en 2018 à ce type de services. Rappelons que cet amendement, comme les dispositions votées en 2018, ne vise qu'à reprendre

D'après les associations de personnes en situation de handicap, tous les travaux visant l'accessibilité des logements ne bénéficient pas d'un taux réduit de TVA, alors même que la directive 2006/112/CE relative au système commun

les ascenseurs ou élévateurs spécialement conçus pour le déplacement de personnes handicapées, pour certains systèmes de douche et de baignoire spécialement conçus pour personnes handicapées, pour des treuils, rampes ou d'autres dispositifs d'accès

pour les immeubles achevés depuis plus de deux ans. Mais, pour ces autres travaux, on est sans doute à la limite des travaux d'amélioration générale du logement. Par ailleurs, M. Savoldelli l'a très honnêtement reconnu, le taux

pas compte. Concernant les aides budgétaires, outre la prestation pour l'aménagement du logement délivrée par les départements, les personnes souhaitant aménager leur logement peuvent, sous condition de ressources, bénéficier des aides de l'ANAH. Cette aide, obtenue sur présentation d'un justificatif de handicap, représente 35 % du montant hors taxes des travaux,

que les contribuables réalisent dans leur habitation principale, au titre, d'une part, des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées, et, d'autre part, au titre des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, dans la limite d'un plafond global pluriannuel de dépenses de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple. Comme vous le savez, le Gouvernement a prorogé la période d'application de ce dispositif au 31 décembre 2020.

aux produits de biocontrôle, tels qu'ils sont définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime. Est ainsi proposée la création d'un nouveau levier fiscal en faveur du développement des produits de biocontrôle. En effet, le déploiement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition d'une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l'agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles, tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse les personnes publiques- État, collectivités territoriales et établissements publics -comme les particuliers, qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1 janvier 2017 pour les unes et du 1 janvier 2019 pour les autres. Dans ce contexte, il est donc essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution, tels que les produits de biocontrôle, qui, en utilisant des mécanismes naturels- organismes vivants ou substances naturelles

Le passage en 2013, puis en 2014, d'un taux réduit de TVA à un taux normal- aujourd'hui de 20 % -a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses pour l'ensemble des acteurs de la filière équine. En janvier 2018, la Commission européenne a proposé de modifier la directive sur la TVA de 2006 en ce qui concerne les taux réduits, pour rendre la main aux États membres et leur permettre de recourir librement aux taux réduits. En France, le taux moyen pondéré varie aujourd'hui autour de 14 %, ce qui offre au Gouvernement une marge certaine. En attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle directive, une révision de l'interprétation de l'actuelle directive sur la TVA s'impose, s'appuyant sur une analyse plus fine de ce qui relève de l'activité sportive, sociale et agricole dans la filière équine et qui, à ce titre, mériterait de bénéficier de nouveau du taux réduit. Le passage au taux normal de TVA pour les centres équestres est peu équitable, car il met en péril une logique de fonctionnement vertueuse : chez nos voisins, les structures équestres sont bien souvent sous modèle associatif, donc non assujetties à la TVA, et les cavaliers possèdent leur propre monture, tandis que notre modèle de cheval partagé rend accessible la pratique de l'équitation sans posséder un cheval. Cependant, depuis 2014, en France, les prestations

équine. Nous sommes déterminés à obtenir une évolution du droit européen, qui prenne en compte les spécificités de ce secteur, dans le cadre des discussions entamées sur la mise en oeuvre du plan d'action sur la TVA, notamment en matière de taux. Nous soutiendrons la possibilité d'appliquer plus largement un taux réduit dans la filière équine. Tel est le cadre de notre

trois quarts de ces entreprises ont connu une augmentation de leurs ventes en 2017, et près de la moitié d'entre elles a connu une croissance à deux chiffres. Parmi les dix premiers groupes mondiaux du luxe,

celle des populations précaires, essentiellement, qui ne fréquentent pas les magasins de luxe, pour des raisons évidentes. Nous proposons de baisser le taux de la TVA à 5,5 % sur les protections périodiques, alors qu'elles étaient jusqu'à présent taxées à 20 %, autant que les produits de luxe. produits de luxe. En 2018, l'Écosse, par exemple, est allée plus loin en distribuant gratuitement ces produits d'hygiène aux écolières et aux étudiantes. Je sais que le Gouvernement envisage une expérimentation : la distribution gratuite des protections hygiéniques dans les écoles, hôpitaux ou prisons, pour lutter contre la précarité menstruelle.

Mme Claudine Lepage. Il y a un an, lors de l'examen du PLF pour 2019, le Sénat a voté l'abaissement du taux de TVA pour les agences de presse de 10 % à 5,5 %. Malheureusement, l'amendement n'a pas été retenu en commission mixte paritaire. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras aujourd'hui. Historiquement, les agences de presse, comme d'ailleurs le livre, bénéficiaient d'un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les cessions d'éléments d'information, et les éditeurs de presse un taux super-réduit de 2,1 %. En 2012, le taux de 5,5 % a été porté à 7 % pour les bénéficiaires de ce taux réduit. Les agences de presse ont accusé le coup. Le 1er janvier 2014, le taux de 7 % a été porté à 10 %, sauf pour le livre, qui a obtenu de revenir à 5,5 %. Quant aux services de presse en ligne, conformément au rapport de la mission menée nous sommes parvenus, à force de dépôts récurrents d'amendements dans les lois de finances successives, à obtenir l'application du taux super-réduit de 2,1 % au 1er février 2014, au lieu du taux normal auquel ils étaient jusqu'alors assujettis. Le manque à gagner pour l'État du passage d'un taux de 10 % à un taux de 5,5 % n'atteindrait même pas 6 millions d'euros. En effet, le passage de la TVA de 5,5 % à 10 % n'a entraîné qu'un bénéfice mineur pour l'État, mais s'est soldé par un appauvrissement des agences de presse et par une nouvelle baisse de leur activité, ce qui, mécaniquement, apporte moins de recettes de TVA dans les caisses de l'État. Dans une économie de coûts fixes, constituée à 75 % de charges de personnel, la dégradation de la trésorerie des agences de presse menace directement l'emploi. Voilà un cercle vicieux extrêmement préjudiciable, qui fragilise des entreprises déjà en difficulté face aux Gafam, qui exploitent jusqu'à maintenant leurs contenus sans les rémunérer, et cela malgré la promulgation de la loi du 24 juillet 2019. Plus que jamais, les agences de presse ont besoin de la solidarité des acteurs politiques et d'un coup de pouce fiscal. Notre amendement vise à rétablir un taux de TVA applicable aux agences de presse à 5,5 %.

Nous estimons que la mesure que vous proposez aurait un impact réduit, en raison du nombre de prestations réalisées entre entreprises assujetties, ayant la possibilité de déduire la TVA. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Quelle incohérence ! D'un côté, vous augmentez la TVA sur les agences de presse, et, de l'autre, au nom du soutien à la diversité, de l'indépendance de l'information et face à la concurrence avec les agences de presse étrangère, l'État est obligé d'accorder

alors qu'il a baissé dans le monde, en particulier en Europe, sous la pression du marché. Comme l'indiquait un article du journal, bon connaisseur de la question, « malgré un taux qui reste élevé aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés rentre mal dans les caisses de l'État ». économiques (OCDE), publiée au début de cette année, indiquait que la France se situait presque en dernière position, si nous considérions la part de l'impôt sur les sociétés dans les recettes fiscales, soit 5 % contre 9 % en moyenne par pays membre de l'OCDE.

qui bénéficie principalement aux détenteurs de capitaux dans les entreprises. Nous proposons, par notre amendement, de maintenir le taux de 33,3 % pour les grosses entreprises, qui doivent participer à la solidarité nationale,

Malheureusement, cet amendement est rigoureusement contraire à la position de la commission, qui regrette justement que le Gouvernement revienne sur ses engagements de baisser de manière pluriannuelle l'impôt sur les sociétés, au moins pour les plus grandes entreprises. L'on nous a déjà fait le coup, et cela recommence ! Hier soir, le ministre Bruno Le Maire nous disait

pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 250 millions d'euros. Il confirme donc la baisse d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises tout en l'atténuant, dans la droite ligne des mesures dites « gilets jaunes » de l'an dernier.

28 % quel que soit le montant du bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2020 ; et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2021. Si la distinction entre les grandes entreprises

De plus, le ministre Bruno Le Maire a estimé que les seuils favorisaient, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, des stratégies d'évitement et d'optimisation. C'est probablement exact

La réalité, c'est que la politique fiscale du Gouvernement en matière d'imposition sur les sociétés est favorable non pas à nos PME, mais plutôt aux grands groupes, et ce n'est pas le taux faiblement différencié actuellement appliqué,

à l'entreprise qui acquiert un équipement numérique de l'utiliser de manière optimale, en maîtrisant pleinement son pilotage et ses différentes fonctionnalités

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs, afin de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d'améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. sont de plus en plus nombreux à s'engager dans la voie d'une production agricole plus respectueuse de l'environnement. Ils doivent être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires qu'ils subissent à répétition, des solutions concrètes doivent leur être proposées. De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l'utilisation de drones en agriculture permettent, d'ores et déjà, de réduire considérablement l'usage des intrants. Se développe, en parallèle, un ensemble de technologies fondées sur l'existence de capteurs permettant, avec des algorithmes qualifiés, de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d'agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu'à 90 %. Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important qu'elles emportent. C'est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d'acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles,

de finances, on nous propose un certain nombre d'aménagements et de suramortissements pour accompagner la transition énergétique.

Il a pour objet d'aligner le régime d'imposition des subventions et des primes d'équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations. Le régime du bénéfice réel permet de payer des impôts sur la base des bénéfices effectivement réalisés. Il soumet les entreprises à des obligations comptables strictes et concerne celles d'entre elles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 80 000 euros pour une activité commerciale. ou du micro-bénéfice agricole, dit « micro-BA », est lui aussi soumis à des obligations comptables souples, la seule contrainte étant la tenue d'un livre de recettes. Il permet, en outre, de bénéficier d'une imposition favorable des subventions au titre du plan Loup. Cette différence de traitement ne semble pas justifiée. C'est pourquoi je vous propose d'adopter cet amendement. Quel est l'avis de la commission ?

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l'article 50 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture placé en deuxième partie. Cette mesure permettra d'avancer au 1 janvier 2020 l'entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue au 1er janvier 2021. L'article 50 sera, en conséquence, supprimé. supprimé. Le présent amendement vise à élargir le champ d'application du mécanisme de paiement étalé de l'impôt sur le revenu de l'article 75-0 C du CGI aux frais de fermage des avances aux cultures et aux charges afférentes aux stocks de produits ou d'animaux dont la valeur a été bloquée, qui, bien qu'ils constituent des éléments incorporables

Cet amendement vise à modifier le montant de l'amende forfaitaire de 1 500 euros, qui avait été introduite par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale et qui vise les sociétés ayant bénéficié, en application de l'article 235 nouveau du code général des impôts, d'une restitution temporaire de retenue à la source du fait de leur situation fiscale déficitaire, mais qui omettent de déposer les documents justifiant de leur droit au maintien de ce report et du quantum de l'imposition toujours Il est donc prévu un montant proportionnel aux enjeux liés au respect des obligations déclaratives des sociétés étrangères concernées. Quel est l'avis de la commission ?

Cet amendement tend à poser la question de la neutralisation fiscale de certains avantages pour les sociétés fiscalement intégrées. Nous considérons que le droit existant ne permet pas d'assurer cette neutralité. Nous avons donc souhaité entendre le Gouvernement,

est défavorable, car le dispositif envisagé revient, de fait, sur la suppression de la neutralisation des subventions et abandon de créances intra-groupe, adoptée l'année dernière, qui avait pour but de mettre le régime de groupe en conformité avec le droit de l'Union européenne. Réserver ce dispositif aux seules entreprises faisant l'objet d'un contrôle n'est pas juste vis-à-vis de celles qui s'efforcent d'appliquer correctement les règles fiscales. En réalité, cela reviendrait à inciter les entreprises à ne pas appliquer la loi. Le dispositif proposé favoriserait les occurrences dans lesquelles la situation financière de la société bénéficiaire lui permet de reverser l'aide intra-groupe, ce qui signifie dès lors que l'aide n'était pas impérative.

clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l'article L. 236-3 du code de commerce, en prévoyant que, en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement détenues par une autre société, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent. Par cette disposition, la fusion ou la scission de sociétés soeurs détenues à 100 % par une même société mère s'effectue sans échange de titres, ce qui paraît assez logique. Le présent amendement vise à procéder aux coordinations nécessaires, afin que le régime fiscal de ces opérations reste comparable à celui des opérations de fusion entre sociétés soeurs donnant lieu à échanges de titres sous l'empire de la législation antérieure au 19 juillet 2019. afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme, cet amendement tend à préciser les conditions d'application du régime du long terme aux plus ou moins-values de cession des titres après réalisation d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres. prévoir les modalités d'appréciation du délai de détention des titres conditionnant l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu au c du 1 de l'article 145 du CGI, lorsque les titres de la société bénéficiaire ou apporteuse sont détenus pendant moins de deux ans après la date de la fusion ou de la scission. Le dispositif proposé s'appliquera rétroactivement à compter de l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 19 juillet 2019 afin que l'ensemble des opérations réalisées dans ce cadre suive le même régime fiscal. Cette mesure vient utilement compléter l'amendement du sénateur Mohamed Soilihi, lequel vise à étendre l'application du régime spécial des fusions et ainsi à assurer la neutralité fiscale des opérations de fusion ou de scission par l'exonération d'impôt sur les sociétés de la plus-value d'apport d'apport dégagée par la société absorbée ou scindée et le sursis d'imposition de cette plus-value pour la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport en cas de scission. Vous l'avez compris, il s'agit d'un amendement technique, qui vise à rendre effectif un dispositif adopté dans la loi du 19 juillet 2019 et à faire en sorte qu'il soit complètement homogène et respecte le principe d'équité fiscale.

à M. Jean-Marie Morisset. Le présent amendement a pour objet de renforcer les seuils permettant d'accéder au régime des sociétés mères, lequel permet la distribution de dividendes en franchise d'impôt dès lors que la société bénéficiaire de la distribution détient 5 % du capital de la société distributrice, voire 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote en cas de dilution. mères non résidentes, ce régime est considéré comme transposant la directive européenne. Si ce régime d'exonération s'est révélé d'une grande stabilité sur le plan interne, il est le support de nombreux contentieux dans le cadre de structures transfrontalières, en particulier au regard de la liberté de circulation des capitaux. En effet, le seuil fixé par l'article 145 est aussi visé, par renvoi, pour l'exonération de la retenue à la source, prévue à l'article 119 du code général des impôts. Alors que le standard européen n'exige d'éliminer la double imposition que pour les détentions en capital supérieures à 10 %, le régime français se révèle plus favorable que la directive, dans la mesure où son bénéfice est ouvert aux sociétés mères détenant entre 5 % et 10 % du capital

et une plus grande lisibilité

disposition l'intéresse au plus haut point, puisqu'elle se rapporte à la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, dont nous avons précédemment parlé. Je suis d'ailleurs surpris que l'examen de l'amendement

extracomptable ; ce système est traditionnellement admis par l'administration fiscale en cas de suppression, par la loi, d'une exonération. C'est pourquoi, dans l'attente des réponses que doit donner l'administration fiscale,

On comprend la volonté de simplification, mais, dans la pratique, ce n'est pas parce qu'un impôt, une taxe, une redevance ou un droit de douane sont mis en recouvrement qu'ils sont effectivement payés.

désaligner obligations comptables et obligations fiscales. Or nous n'avons pas connaissance, mais peut-être simplement faute d'informations, de difficultés particulières dans l'application de ces principes.

de résultats d'exploitation soumis tout à la fois à l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif et aux cotisations sociales personnelles, les entreprises concernées voient leurs capacités d'autofinancement considérablement réduites. Sans attendre le lancement d'une réflexion sur les aménagements à apporter au statut des entreprises individuelles et des sociétés relevant du régime de l'impôt sur le revenu, une mesure autorisant ces entreprises à constituer une provision pour investissement serait, dans l'immédiat, de nature à débloquer de nombreux projets indispensables à leur croissance. Quel est l'avis de la commission

-et, sur délibération des collectivités territoriales, d'exonérations d'impôts directs locaux. Ce dispositif comprend, en outre, un volet social, consistant en une exonération de cotisations sociales patronales s'appliquant durant les huit années suivant la création de l'entreprise, quelle que soit la date à laquelle cette création est intervenue. intervenue. L'efficacité du dispositif des JEI, très ancien et qui a traversé les différentes législatures, est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d'incitation fiscale aux activités de recherche et développement, au sein des vingt-six États membres de l'Union, et cette étude classe notre dispositif de soutien en première position, à l'échelle européenne. Nous voulons donc vraiment le maintenir et lui donner toute sa force. Afin de donner la visibilité adéquate aux créateurs d'entreprises innovantes, le présent amendement tend à proroger ce dispositif d'exonérations fiscales jusqu'au 31 décembre 2022. Cette mesure n'emporte pas de conséquence sur le dispositif d'exonération sociale, puisque celle-ci n'est actuellement soumise à aucun bornage temporel. Par ailleurs, l'obtention du statut de JEI est actuellement subordonnée à la réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'entreprise. Or la volatilité des cours, tant en monnaies étrangères qu'en cryptomonnaies, ainsi que la volatilité du marché des valeurs mobilières de placement, notamment sur ce type d'entreprises, peuvent conduire à la constatation de pertes latentes et de moins-values, pour des raisons totalement indépendantes

Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l'activité, mais il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun. C'est pourquoi le présent amendement vise à limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d'être soumis au régime de la micro-entreprise. En effet, la législation actuelle a conduit à des distorsions inacceptables de concurrence entre l'entrepreneur qui exerce en nom propre, dans le cadre d'un régime de droit commun, et celui qui opte pour le régime de la micro-entreprise. Par ailleurs, dans le cadre du grand débat national, nombre de chefs d'entreprise de proximité se sont exprimés sur cette question, dénonçant le fait que, un devis présente, dans un cas, un surcoût de TVA et, dans l'autre, non. L'équité élémentaire exige que, pour la même activité exercée, les entrepreneurs acquittent les mêmes charges, quels que soient le statut ou le régime fiscal ou social de l'entreprise.

Le présent amendement vise à accompagner les apiculteurs ayant plus de cinquante ruches, en appliquant l'imposition à partir de la cinquante et unième. En exonérant d'impôts les cinquante premières ruches, il s'agit d'aider les apiculteurs à faire face aux importantes pertes annuelles de cheptel, qui nécessitent de renouveler, chaque année, les investissements.

qui est assez favorable et qui a harmonisé les règles de détermination du bénéfice pour les petits exploitants agricoles en règle générale. Il ne nous semble pas souhaitable d'y revenir en créant des exceptions

Le dispositif de l'épargne de précaution porté à l'article 51 de la loi de finances pour 2019 a créé un nouveau levier stratégique essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques. Afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d'utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, notre collègue Daniel Gremillet propose d'adapter l'épargne de précaution aux spécificités de l'agriculture de groupe. À cette fin, il propose de modifier le dernier alinéa de l'article 73 du code général des impôts. Quel est l'avis de la commission ?

Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux de tenir une comptabilité propre à ces activités, en sus de la comptabilité liée à leur activité agricole. Il est proposé, à titre de règle pratique, d'appliquer au résultat de l'exploitant, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice, puis d'exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles, ou d'imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux. Ce rapport, aisé à déterminer par l'exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 75 du code général des impôts. Il s'agit d'une mesure de clarification et de simplification. La

Assurant la formation de leurs membres à la comptabilité, les assistant dans l'établissement de leurs déclarations annuelles, les amenant, le cas échéant, à corriger certaines erreurs, ces organismes ont pleinement rempli les missions qui leur ont été confiées. En contrepartie des sujétions particulières liées à leur adhésion, leurs membres se sont vu accorder un avantage prenant la forme d'un abattement sur leur bénéfice imposable. imposable. Cet équilibre initial a été gravement mis à mal par deux vagues de réformes récentes. D'une part, l'avantage positif lié à l'adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a été supprimé et remplacé par un « avantage » négatif : celui qui n'adhère pas à un organisme agréé se voit pénalisé par une imposition calculée sur un bénéfice rehaussé de 25 %. D'autre part, depuis une réforme intervenue voilà quatre ans, les adhérents d'un organisme de gestion agréé se voient désormais soumis à des « examens périodiques de sincérité » consistant à rapprocher pièces justificatives et écritures comptables, ce qui présente toutes les caractéristiques d'une vérification de comptabilité.

d'organismes de gestion agréés tout en conservant à ces mêmes organismes l'ensemble de leurs prérogatives. En contrepartie des contraintes liées à l'adhésion, les entrepreneurs qui accepteraient d'adhérer à un organisme de gestion agréé bénéficieraient d'un abattement de 10 % sur leurs bénéfices imposables. Quel est l'avis de la commission

L'Inspection générale des finances a finalisé son rapport, qui est en cours de présentation dans les administrations. Nous sommes également en contact avec

Une étude récente a montré que 40 % des profits de ces sociétés échappaient à l'impôt, pour l'essentiel grâce à des transferts artificiels en direction des paradis fiscaux. Le principe de l'amendement est simple : les multinationales, qu'elles soient actives dans le secteur du numérique ou non, doivent payer leur impôt là où elles réalisent leur activité. Ces multinationales masquent leurs bénéfices réalisés en France

dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou le Canada, où un impôt sur les sociétés peut aussi être perçu à l'échelon local. L'État de Californie a ainsi établi son propre impôt sur les sociétés à un taux d'environ 10 qui s'ajoute à l'impôt fédéral sur les sociétés, désormais fixé à 21 %. Si Coca-Cola réalise 10 % de ses ventes en Californie, alors 10 % de ses profits sont taxables dans cet État. Quel est l'avis de la commission ?

Cette avancée notable reste réservée aux entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition, excluant de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d'imposition sur les sociétés. Or ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face. Alors que les entreprises agricoles sont encouragées à choisir l'imposition sur les sociétés, il apparaît contradictoire d'empêcher celles d'entre elles qui font ce choix d'utiliser le dispositif d'épargne de précaution.

Éric Bocquet. Il vise à créer la notion d'établissement stable pour les entreprises ayant une présence numérique significative en France.

d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2022, sous certaines conditions, et notamment sous condition d'un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements. L'amendement vise à préciser que, en cas de fusion, l'engagement souscrit par l'organisme absorbé n'est pas rompu lorsque l'organisme absorbant s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à l'organisme absorbé pour le respect de l'engagement dans le délai restant à courir.

de locaux commerciaux, à condition qu'ils réinvestissent les sommes correspondantes dans les quatre ans dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux. En réalité, cet amendement vise à réactiver un dispositif qui s'était appliqué entre 2006 et 2010.

viticole. La constitution de stocks est un élément de l'activité des entreprises qui engendre des charges financières importantes : des immobilisations financières liées à la conservation du produit, de quatre à cinq en Champagne par exemple, voire de huit à neuf ans dans la région délimitée Cognac. En moyenne, ces stocks, qui représentent plus de trois années de chiffre d'affaires, ont une incidence importante sur le compte d'exploitation des entreprises. Ils nécessitent des immobilisations en bâtiments et matériels pour assurer le stockage et la conservation de ces produits, des charges de personnel supplémentaires liées aux travaux spécifiques d'élaboration et de manutention des produits stockés. La constitution de stocks permet donc d'amplifier la création de valeur sur ces vins élaborés dans les terroirs viticoles français, lesquels contribuent très fortement à la balance commerciale de la France, et elle en a bien besoin. La loi de finances pour 2013 avait procédé à la réintégration, dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, des charges financières nettes à hauteur de 25 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise était supérieur à 3 millions d'euros. Une exception à cette disposition avait été introduite, qui excluait de la base des charges financières nettes soumises au plafonnement de déductibilité les charges financières afférentes aux contrats de financement de stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. ans. Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et a ainsi supprimé cette exception relative au financement des stocks à rotation lente. Les entreprises concernées réalisent de lourds investissements sur les marchés d'exportation pour faire connaître leurs produits. Ils ouvrent également de nouveaux marchés au bénéfice de la filière tout entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et réduit leurs investissements, à un moment où l'avenir de la filière passe par la conquête de nouveaux marchés où les investissements dans la distribution sont d'autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents, pour citer le champagne, n'y est pas habituelle. Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l'ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants. Enfin, les entreprises capables d'exporter sont celles qui atteignent une certaine taille. Leur chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros et leurs besoins de financement sont supérieurs à 100 millions d'euros. Pour préserver leur capacité d'investissement sur les marchés à l'export, il est donc indispensable d'exclure de nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et au stockage.

car nous en avons discuté de manière informelle avec la Commission européenne. Le Gouvernement ne peut pas prendre le risque avéré d'une procédure d'infraction pour mauvaise transposition de la directive. Je le souligne, l'exception qui existait pour les concessionnaires et les délégataires de service public a pu être maintenue, car elle a été prévue dans la directive

Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les SPL ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d'égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité, alors qu'elles ont pour objet la gestion d'un service public. C'est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, tend à prévoir une évolution de l'article 238 du code général des impôts, afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Afin de ne pas dénaturer l'esprit de ce dispositif, l'éligibilité des sociétés de capitaux a été strictement limitée. Les collectivités locales n'ont pas l'obligation de créer des sociétés publiques locales pour mener à bien leurs missions. Le Gouvernement n'entend pas étendre le champ des activités éligibles à la réduction d'impôt.

j'ai été sollicité par la Maison des artistes pour déposer un amendement visant à modifier l'article 238 AB du code général des impôts relatif aux dépenses d'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants ou d'instruments de musique effectuées par des entreprises. projet de loi de finances pour 2019, les sommes relatives aux acquisitions d'oeuvres originales d'artistes vivants sont déductibles de l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise, dans la limite de 10 000 euros ou 5 pour mille de son chiffre d'affaires, lorsque ce dernier montant est plus élevé. telle évolution législative fait suite à plusieurs rapports parlementaires appelant à une modification de l'outil fiscal relatif au mécénat et à l'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants, notamment au profit des plus petites entreprises. s'agissant de l'art contemporain, le montant annuel de déduction reste anormalement limité. En effet, la déduction obtenue au titre des dépenses d'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants est d'abord diminuée des réductions d'impôt dont l'entreprise aura par ailleurs pu bénéficier au titre de ses dépenses de mécénat. Ensuite, si ces dépenses sont déductibles du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, le montant n'ayant pu être déduit au cours de l'exercice « n » ne peut être reporté. Il est donc définitivement perdu. le dispositif actuel prévu par l'article 238 AB réduit techniquement à un niveau très bas le plafond de déduction relatif à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants.

présentés. Pour répondre à cette situation, le présent amendement vise à aligner le plafond de déduction annuelle des dépenses d'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants sur celui du mécénat. Il a également pour objet de supprimer, pour le calcul du plafond de déduction des dépenses d'oeuvres d'art, la prise en compte du montant des dépenses de mécénat effectuées au cours de l'année. cet amendement doit permettre aux entreprises de ne pas avoir à choisir entre leur engagement en faveur du mécénat et le soutien à l'art contemporain, en raison du plafonnement global des deux catégories de dépenses. Quel